est pourtant le quotidien de milliers de familles, de mères, d’enfants et de nourrissons, contraints de survivre dans la rue, enchaînant des solutions d’hébergement précaires, temporaires et inadaptées. Dans le XVIII arrondissement de Paris, dont je suis l’élu, le centre d’hébergement Suzanne Valadon accueille des familles en détresse. Je m’y suis rendu dimanche dernier pour rencontrer ces familles – mères et enfants – qui, après des mois d’errance, y ont trouvé un toit. Mais il s’agit d’un toit temporaire. Derrière les chiffres, il y a des visages et des regards d’enfants. Il y a Pierre Maël, âgé de 5 ans, qui se réveille chaque nuit en pleurant, car sa chambre est infestée de souris. Pour lui, la nuit est non pas un moment de repos, mais une source d’angoisse. Il y a encore la petite Anne Laure, âgée de 3 ans, qui n’a jamais connu la stabilité, et ignore ce qu’est un foyer sûr et durable. Ces enfants, comme tant d’autres, ne vivent pas : ils survivent. Certains ont trouvé refuge dans des gymnases, des urgences hospitalières, des églises. D’autres dorment dans la rue, dans des abris de fortune, dans des chambres d’hôtel parfois miteuses ou des squats. Nourrissons, enfants en bas âge, adolescents : tous sont exposés à l’insécurité et à une précarité extrême. Cette situation – nous en sommes, je le pense, collectivement convaincus – n’est ni une fatalité ni une conséquence inévitable des crises économiques. Elle est le résultat d’un manque de décisions politiques et économiques, d’une absence de volonté réelle de faire du droit au logement une priorité nationale. Nous avons aujourd’hui l’occasion d’envoyer un message fort : nous ne tolérons plus que des enfants dorment dehors. La France aime, à juste titre, se présenter comme le pays des droits de l’homme. Nous sommes d’ailleurs signataires de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) depuis 1989. Nous la citons dans les débats internationaux, nous nous en réclamons

Cet engagement fait peser sur l’État, sur nous, une obligation claire, celle de garantir aux enfants un cadre de vie stable et sécurisé. L’ONU a d’ailleurs rappelé cette exigence au travers de l’observation générale n° 21 du Comité des droits de l’enfant, qui souligne la vulnérabilité des enfants vivant dans la rue et l’impératif pour les États de mettre en place des politiques publiques adaptées et pérennes afin de faire Nous ne sommes clairement pas à la hauteur de ces engagements. Le dire n’est pas mettre en cause tel ou tel gouvernement, tel ou tel ministre, car force est de constater qu’il s’agit d’un échec global. Nous ne pouvons pas nous contenter d’afficher de grands principes si, dans la réalité, nous ne garantissons pas ces droits fondamentaux aux enfants de notre pays. Car les chiffres que nous avons sous les yeux sont alarmants. Le 19 août 2024, l’Unicef et la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS) ont recensé plus de 2 000 enfants sans solution d’hébergement. Ce chiffre a plus que doublé en trois ans. Parmi eux, 467 enfants avaient moins de 3 ans. À Paris, ce sont environ 400 enfants qui dorment dehors. Dans la métropole de Lyon, ils étaient plus de 300 à la fin de l’année 2023, soit une augmentation de 40 % en un an et de plus de 200 % en deux ans, selon le collectif Jamais sans toit. Derrière ces chiffres, il y a des visages, des vies qui, souvent très jeunes, sont exposées à une extrême précarité. Concrètement, cela signifie que des centaines de nourrissons et d’enfants dorment chaque soir dans la rue, sans protection, exposés à tous les dangers. Ces chiffres ne sont que la partie émergée de l’iceberg. Ils ne prennent pas en compte les familles qui ne sollicitent plus le 115, lassées d’attendre un hébergement qui ne vient pas. Ces enfants sont sans repères et sans protection. Ils grandissent dans la peur, l’incertitude et l’indignité. C’est la raison pour laquelle il est nécessaire de prendre en compte l’ensemble des conséquences du sans abrisme des enfants. Nous savons que le fait de vivre à la rue, même temporairement, laisse des séquelles profondes : troubles du sommeil, anxiété, stress post traumatique – la liste est bien longue… Le mal logement, quant à lui, multiplie par 1,5 le risque de retard scolaire. Il a un coût pour l’État en raison des redoublements qu’il engendre. Il est de notre responsabilité d’agir

Considérer que des enfants peuvent continuer à dormir dehors, c’est renoncer à notre propre humanité. Sur un tel sujet, nous avons besoin, à l’évidence, de dépasser les clivages politiques traditionnels, de nous rassembler, de nous unir autour d’un seul et même objectif : faire en sorte qu’il n’y ait plus d’enfant qui dorme à la rue.

des hommes et des femmes désireux de s’engager en vue de mettre fin à l’extrême pauvreté. En 1991, interrogée sur le sens de cet engagement qui se poursuivra pendant plus de trente ans, Geneviève de Gaulle Anthonioz déclarait Quand j’ai découvert que les droits de l’homme, dans mon propre pays, après qu’on ait combattu pour ça, n’étaient pas respectés, parce que la misère ce n’est pas les droits de l’homme, ça m’a fait un drôle de choc. » Ce choc est encore le nôtre aujourd’hui, je suis heureux que cette proposition de résolution transpartisane visant à mettre fin au sans abrisme des enfants nous permette, d’une part, d’appeler le Gouvernement

pas par de bons résultats : sur le sujet du mal logement, la France accuse un retard. Si la question du sans abrisme des enfants est au cœur de nos préoccupations aujourd’hui, je voudrais commencer par rappeler que c’est l’état du mal logement dans son ensemble en France qui est préoccupant. Au moins 4,2 millions de nos compatriotes sont mal logés, logés, dont 350 000 sont sans domicile. Les 3,85 millions de personnes restantes vivent, pour les unes, dans des abris de fortune, pour les autres, dans des taudis ou dans des logements surpeuplés. Les plus chanceux auront réussi à trouver une place en structure d’accueil ou en hébergement temporaire à l’hôtel, dans les conditions décrites par Ian Brossat. Nous ne saurions nous habituer à cette situation indigne du grand pays qu’est la France, indigne pour tout homme quel qu’il soit et d’où qu’il vienne. Cette réalité, ce choc auquel nous devons nous confronter, n’est pas une nouveauté. Au contraire, elle s’aggrave et appelle à un réveil collectif entre 2012 et 2014, le nombre de personnes sans domicile a augmenté de 145 %. L’incapacité à trouver des places d’hébergement d’urgence pour ces femmes et ces hommes explique en partie cette croissance préoccupante. Certes, nous ne sommes pas restés totalement inactifs, l’augmentation du nombre de places d’hébergement de 150 000 en 2017 à 200 000 en 2023 en témoigne. en 2023 en témoigne. Mais sur cette question nous ne saurions nous réjouir d’un résultat partiel. Concrètement, il nous faut financer nos ambitions. Sur ce plan, on constate une surexécution chronique du programme 177 Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables » de nos lois de finances. Cette surexécution se chiffre à un montant annuel proche d’environ 200 millions d’euros. La sous budgétisation d’un programme clé prive les opérateurs de la mission de la possibilité de mener sereinement leurs actions. Alors que le stock de places n’a cessé de croître, qu’attend on pour pérenniser un financement cohérent avec les besoins ? Certaines associations font ainsi part des difficultés liées à ces incohérences. Les surcoûts liés à la fermeture puis à la réouverture de places s’accompagnent d’un manque grave d’efficacité qu’il nous faut pallier. De même, des actions au profit des personnes hébergées ne donnent parfois lieu au décaissement des crédits que tardivement, voire après leur réalisation, ce qui peut mettre en péril les plus petites structures. Soyons au rendez vous aux côtés de ceux qui s’engagent concrètement pour soutenir les plus démunis. Au cœur de cette réalité tragique se situe la question qui nous réunit aujourd’hui : celle, peut être plus tragique encore, du sans abrisme des enfants. Ici encore, le choc éprouvé par Geneviève de Gaulle Anthonioz, que j’évoquais au début de ma prise de parole,

par rapport à 2020 et, parmi ces 2 000 enfants, 467 ont moins de 3 ans. Pourquoi ceux ci ont ils passé la nuit du 19 août 2024 dehors ? Parce qu’ils se sont vu opposer une impossibilité d’être pris en charge. Là encore, l’on aurait aimé pouvoir se rassurer en se disant que la France, patrie des droits de l’homme, était à la pointe de la lutte contre la pauvreté touchant les enfants. Mais non, car en Europe, la France fait, une fois de plus, figure de mauvais élève. La lecture du neuvième Regard sur le mal logement en Europe publié par la Fondation pour le logement des défavorisés est, à ce titre, édifiante. L’on y apprend que, dans notre pays, plus de 25 % des mineurs sont en risque de pauvreté ou d’exclusion sociale. C’est le sixième taux le plus haut de l’Union européenne. Pire encore : en France, la part de ménages avec enfants vivant sous le seuil de pauvreté dans un logement insalubre a augmenté de plus de 40 %. Cela nous classe à l’avant dernière place sur vingt sept. Nous ne pouvons tolérer que, dans notre pays, en 2025, des enfants puissent encore rencontrer ce genre de difficultés. Trop souvent invisibilisées, nous pensons que ces réalités appartiennent à un temps révolu, or elles sont pourtant bien là et elles nous appellent à agir. Certes, ici encore, des progrès ont été réalisés : la loi de finances pour 2025 retient l’ouverture de 1 000 places pour les enfants dans le parc d’hébergement d’urgence, ainsi que 1 000 places pour les femmes proches de la maternité.

de mieux considérer le cas des femmes avec enfants dans le cadre de l’hébergement d’urgence en assurant à ces dernières davantage de places adaptées à leur configuration familiale, notamment en vue de leur permettre de disposer de plus d’intimité. En second lieu, n’oublions pas le travail remarquable réalisé par les travailleurs sociaux dans notre pays : leur profession et leur statut méritent d’être revalorisés. Enfin, je tiens à rappeler que la gestion de l’urgence ne saurait être une fin en soi. Car, pour les enfants sans abri, ce qui manque est non pas seulement le toit, mais l’accès à l’ensemble de leurs droits : l’école, évidemment, mais aussi la santé, physique comme mentale. J’appelle le Gouvernement à agir pour permettre à ces enfants et à leurs familles d’être réintégrés au mieux et au plus vite. Cela passe, notamment, par un accès à des logements pérennes à bas prix. Mes chers collègues, les défis que notre pays rencontre actuellement sont immenses, sur le plan tant national qu’international. Mais ne commettons pas l’erreur d’oublier à cette occasion les plus vulnérables d’entre nous. La parole

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la proposition de résolution transpartisane que nous examinons aujourd’hui est, sans aucun doute, révélatrice de la situation sociale que nous connaissons actuellement. C’est aussi le signe d’une insuffisance des politiques publiques pour répondre à une évolution inquiétante du sans abrisme. Je ne peux que remercier vivement notre collègue Cécile Cukierman pour cette initiative qui permettra de mettre des mots sur ces situations que nous croisons tous les jours sans vraiment y prêter attention, de mettre des mots sur ces souffrances que nous tendons à banaliser, de mettre des mots sur l’indicible.

victimes d’une invisibilisation parfois volontaire pour ne pas s’exposer aux violences de la rue. Elles seraient près de 120 000 dans nos rues. Certes, la majorité d’entre elles bénéficient d’un hébergement financé par l’État. Mais il reste celles qui n’ont comme seul toit que le ciel, parfois étoilé. Leurs enfants les accompagnent souvent. Près de 3 000 d’entre eux partagent la précarité de leurs parents chaque soir, dans nos rues. Nous ne pouvons accepter que des enfants grandissent dans l’incertitude, la précarité et sans un foyer stable. Chaque jour passé dans la rue est un jour volé à leur enfance et à leur avenir. Nous ne pouvons nier les répercussions sur leur santé physique et mentale, leur développement ou encore leur scolarité. Aucun enfant ne mérite de vivre un tel traumatisme. En tant que mère de famille, je resterai à jamais marquée par certaines rencontres lors des maraudes auxquelles je participe avec l’Ordre de Malte. Je revois régulièrement ces yeux d’enfants rougis par la faim, ces têtes abaissées par la honte. Mais je garde en moi, comme de précieux souvenirs, ces sourires innocents et ces gestes de reconnaissance. Ils nous rappellent l’importance d’agir. Mes chers collègues, je vous invite à nous rejoindre au sein de la Maraude des parlementaires. Offrir trois heures de notre temps peut être plus bénéfique, plus fort, que de longs discours. Les mots passent, le mal logement et le sans abrisme demeurent et gagnent même en ampleur. Par expérience, nous savons que personne ne peut détenir la solution. En 2022, le Gouvernement s’était engagé à ce qu’aucun enfant ne dorme à la rue.

En l’espace de dix ans, le Gouvernement a triplé les crédits consacrés à sa politique d’hébergement des sans abri. La Cour des comptes a estimé que la stratégie retenue appréhendait surtout les besoins en matière d’hébergement d’urgence comme étant temporaires. Force est de le constater, ces besoins perdurent et s’amplifient avec le temps. L’initiative de notre collègue Cécile Cukierman a le mérite de ramener cette question au centre du débat. Permettez moi d’exprimer au moins un regret. Une grande partie du sans abrisme chez les enfants est liée à des situations familiales précaires. Il est donc crucial de soutenir les familles, de leur offrir un accompagnement social

comme bénéficiaires directs de l’accompagnement psychosocial global destiné aux parents. De même, nous estimons crucial de renforcer les moyens alloués aux dispositifs de médiation scolaire, en particulier pour garantir l’inscription des enfants à l’école sans exiger un justificatif de domicile. Nous partageons tous sur ces travées un même constat et une même ambition : mettre fin au sans abrisme des enfants ne peut être un objectif ponctuel, cela doit être une priorité constante de tous, avec des moyens à la hauteur de l’enjeu. Au sein du groupe RDPI, nous partageons pleinement l’objectif de cette proposition de résolution. Nous sommes convaincus qu’elle représente une étape décisive dans l’engagement que nous devons aux enfants les plus vulnérables, mais cette étape n’est pas une fin en soi. Le vote de cette proposition de résolution confirmera notre volonté de lutter efficacement

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues,

Cosigné par des sénateurs issus des huit groupes, il témoigne d’une prise de conscience partagée au sein de notre assemblée. Le RDSE est particulièrement sensible à la protection des enfants. C’est dans cet esprit que nous avions fait adopter la proposition de loi loi renforçant la protection judiciaire de l’enfant victime de violences intrafamiliales. La situation que nous évoquons aujourd’hui est d’une gravité extrême. La question du sans abrisme des enfants relève non pas d’un simple enjeu social ou budgétaire, mais bien de la dignité, des droits fondamentaux et du respect du contrat républicain. Nelson Mandela disait : « Rien ne révèle mieux l’âme d’une société que la façon dont elle traite ses enfants. » Forts de cette conviction, nous devons agir avec détermination. Selon un baromètre réalisé par Unicef France et la Fédération des acteurs de la solidarité, plus de 2 000 enfants se sont retrouvés sans solution d’hébergement à la fin du mois d’août dernier. Au total, plus de 6 700 personnes n’ont pas trouvé de place en hébergement d’urgence. Cette saturation du dispositif témoigne d’un manque criant de solutions adaptées. Derrière ces chiffres, il y a bien sûr des vies, notamment celles des enfants dont le quotidien est marqué par l’incertitude et la peur. Nous savons combien l’absence de logement stable peut être dévastatrice. D’après une étude menée par Unicef France et le Samu social de Paris, un enfant sans domicile a deux fois plus de risques de développer des troubles de la santé mentale. Comment grandir, apprendre et se construire un avenir quand on vit dans de telles conditions ? Que dire également des 28 000 enfants qui vivent à l’hôtel, privés du cadre stable dont ils ont besoin pour grandir dignement ? Ce mode d’hébergement est non seulement coûteux, mais aussi totalement inadapté. Comment peut on espérer qu’un enfant s’épanouisse dans un environnement aussi précaire ? Il est indispensable de privilégier des solutions de logement plus durables et mieux adaptées à la vie familiale et au développement de l’enfant. Rappelons le avec force : aucun enfant ne doit dormir dans la rue ! C’est une évidence. Pourtant, malgré les engagements répétés des gouvernements successifs, la promesse n’a pas été tenue. Certes, des efforts ont été faits, portant la capacité d’hébergement à 203 000 places. Mais cela reste insuffisant face à l’ampleur des besoins. Madame la ministre, nous connaissons votre engagement dans la lutte contre le sans abrisme. Mais comment aller plus loin ? L’effort doit être amplifié, car les défis à relever sont immenses. Les logiques de gestion de crise et d’urgence doivent être dépassées. La précarité n’est pas une fatalité. Des solutions existent. Le plan Logement d’abord et le pacte des solidarités constituent des avancées, certes, mais ce n’est pas suffisant. Un des outils essentiels dans cette lutte est l’observatoire du sans abrisme, qui doit nous permettre d’évaluer précisément les besoins et d’orienter efficacement les politiques publiques. Pourtant, cet observatoire peine à fonctionner pleinement, ce qui limite notre capacité à répondre aux besoins des plus vulnérables. Sa relance est une nécessité absolue. Au delà du logement, c’est tout un accompagnement global qui doit être repensé. Le Comité des droits de l’enfant des Nations unies l’a rappelé l’accès à l’éducation, aux soins, à la stabilité sociale de ces enfants doit être une priorité. Il est ici question de leur avenir : c’est aussi un enjeu de société. Pour toutes ces raisons, les sénateurs du groupe du RDSE voteront unanimement ce texte. Nous refusons de détourner le regard.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, lors des débats budgétaires, j’ai été rapporteur pour avis, au nom de la commission des affaires sociales, du programme 177 « Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables ». Dans le cadre de ces travaux, j’ai découvert les chiffres effrayants de la souffrance dans la rue, aujourd’hui, en France.

Le système est totalement saturé. Parmi les familles hébergées, on note une surreprésentation des familles monoparentales, ainsi qu’une forte proportion d’enfants en bas âge, puisque 29 % des enfants Au sein du parc d’hébergement d’urgence, en août 2024, 75 % des personnes accueillies appartenaient à des familles. Pourtant, l’hôtel est un lieu inadapté au développement des enfants. Il ne permet pas à ces derniers d’acquérir une autonomie, d’avoir une vie affective ou de bénéficier d’un lieu calme pour poursuivre une scolarité. De plus, selon le Samu social de Paris, 40 % des personnes hébergées en hôtel ne mangent pas à leur faim. Ces chiffres ne tiennent pas compte des familles sans solution d’hébergement après un appel au 115, alors que 59 % des demandes non pourvues concernaient des personnes avec enfants,

ou par peur de se voir retirer leurs enfants, ne sont pas comptabilisées, non plus que les mineurs non accompagnés (MNA) en situation de rue, qui sont pourtant des enfants. Face à ce constat dramatique, plusieurs remarques si l’on doit distinguer les enfants effectivement dans la rue de ceux qui bénéficient d’un toit temporaire, il faut cependant considérer que tous sont en danger. Deuxièmement, le programme « Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables » manque d’efficience, et une prise en charge en hébergement d’urgence n’a rien d’un parcours d’insertion. Troisièmement, les enfants ne sont pas des statistiques, et chacun d’eux devrait pouvoir écrire son histoire de vie dans des conditions sereines. Sur les dangers que courent les enfants sans abri ou sans domicile, le bilan est sans appel. Le logement est un facteur environnemental central, et le fait d’en être privé le confronte à des conditions de vie dégradées.

D’autres bénéficient d’hébergement d’urgence, parfois dans le long terme, parfois avec des rotations et des retours à la rue. Beaucoup intériorisent leur trouble. L’un d’eux témoigne : « Je me sens étouffé, j’ai pas beaucoup d’espace pour dépenser mon énergie, donc je suis vite en colère. Alors que la Convention internationale des droits de l’enfant reconnaît à chacun d’eux, sans distinction aucune, le droit de jouir du meilleur état de santé possible, la santé mentale des enfants sans domicile est systématiquement compromise dès le plus jeune âge. Ces enfants connaissent des réalités très différentes, mais sont tous confrontés à une précarité multidimensionnelle, qui touche à leurs conditions de vie, économique, sociale et administrative. Les études montrent que les enfants sans abri en âge d’être scolarisés sont deux fois plus susceptibles de souffrir de problèmes de santé mentale que les enfants logés de familles Face à ce phénomène dramatique que l’on ne peut feindre d’ignorer, je dois souligner le maintien dans le projet de loi de finances pour 2025 à un niveau budgétaire constant du programme 177, garantissant ainsi 203 000 places d’hébergement d’urgence. cependant dénoncer une sous budgétisation chronique de ce programme, qui ne correspond non pas à une dérive des dépenses, mais au report d’un déficit ancien. Ainsi, chaque année, il manque 250 millions d’euros à la programmation initiale du budget 177. C’est une forme d’insincérité, qui place les opérateurs du sans abrisme dans une situation d’insécurité et de risque. Si, en décembre 2023 et en décembre 2024 – je sais que vous y avez travaillé, madame la ministre –, les 250 millions d’euros manquants ont pu finalement être affectés aux comptes de fin de gestion, il n’en reste pas moins que les associations ont annoncé ne plus pouvoir fonctionner avec un règlement incertain et des prestations fournies. Leurs trésoreries sont mises à mal. Elles ne peuvent pas optimiser le nombre de nuitées achetées, en les mutualisant dès le début de l’année. Un grand nombre d’entre elles risquent de disparaître et, avec elles, le dernier filet de sécurité des politiques publiques, au plus près des plus fragiles. Si une politique volontariste doit être menée sur le volet du logement, le soutien des acteurs associatifs doit par ailleurs rester une priorité. Le mot progrès n’aura aucun sens tant qu’il y aura des enfants malheureux », disait Albert Einstein. Il est douloureux de penser aux enfants sous les bombes, tués ou brisés par les horreurs de guerres qu’ils ne comprennent pas, aux enfants qui meurent de faim ou de soif sur des terres arides et stériles, aux enfants chahutés par des adultes sans scrupules qui, d’une manière ou d’une autre, ne les respectent pas, aux enfants malheureux d’ici ou d’ailleurs, qui quittent trop vite le temps sacré de l’enfance. N’oublions pas ces petits invisibles dans la rue ou dans les hôtels sordides, nos voisins,

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune. » Nous connaissons toutes et tous ces phrases : elles forment l’article 1 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, écrite il y a près de deux

Cette nuit là, 5 835 personnes n’avaient pas pu obtenir de place d’hébergement d’urgence par le 115 ; 1 728 enfants en faisaient partie, et 379 d’entre eux avaient moins de 3 ans. Cette nuit là, à Paris, il faisait 4 degrés. Un autre chiffre nous accable : en 2024, 735 personnes sont mortes à la rue. La plus jeune avait 2 mois. Ce sont

Ce texte renforce la peur de toutes ces familles, qui doivent partir d’elles mêmes ou risquer des amendes supplémentaires, et les expose à la violence physique et psychologique d’une possible intervention policière. En vingt ans, le nombre d’expulsions locatives a augmenté de 150 %. Derrière ces chiffres, il y a des personnes qui méritent d’avoir un toit. France, septième puissance mondiale, doit pouvoir proposer un hébergement, et même un logement, à ces personnes, selon leurs ressources, y compris quand elles n’en ont aucune. Laisser cette misère perdurer, c’est déshumaniser nos concitoyennes et nos concitoyens qui en souffrent, mais c’est aussi perdre nous mêmes une large part de notre humanité.

Je ne veux plus, d’ici la fin de l’année, avoir des femmes et des hommes dans les rues, dans les bois ou perdus. » Ces mots d’Emmanuel Macron datent de juillet 2017. Depuis, nous comptons 330 000 personnes sans domicile fixe, un chiffre qui aurait dû tomber à zéro en 2017, mais qui a finalement doublé en dix ans. Les 210 000 places d’hébergement ne suffisent donc pas, loin de là.

d’agir. Ensuite, dès le 31 mars, fin de la trêve hivernale, et le 15 avril, fin de la trêve cyclonique à La Réunion, empêchons les expulsions sans solution de relogement, particulièrement lorsque des enfants sont concernés. Votons, lors du budget, les crédits nécessaires pour permettre à tous les enfants d’être mis à l’abri. Travaillons à construire davantage de logements accessibles au plus grand nombre, accessibles à tout le monde, en encadrant mieux les loyers. Le logement doit être un droit, peut être le premier de tous, qui ne peut être confié à un marché

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, permettez moi d’abord de saluer le travail de nos camarades communistes Cécile Cukierman et Ian Brossat pour leur excellente initiative, essentielle et même vitale pour notre cohésion sociale.

Cette phrase de Nelson Mandela résonne avec une acuité particulière lorsque nous regardons la réalité insupportable du sans abrisme infantile en France. Aujourd’hui, dans la sixième puissance économique mondiale, plus de 2 800 enfants les représentants de l’Unicef, avec lesquels j’échangeais encore ce matin – dorment dans la rue faute de solution d’hébergement. Parmi eux, 25 % ont moins de 3 ans. Ces chiffres, en constante augmentation, traduisent l’échec d’une politique publique incapable d’assurer un droit fondamental : celui d’avoir un toit. Derrière ces statistiques glaçantes se cachent des visages, des destins brisés et des enfances sacrifiées. Chaque nuit, des centaines de familles confrontées à l’exclusion sociale doivent affronter l’insécurité, le froid et la peur. Les conséquences sur les enfants sont dramatiques : perturbations scolaires, troubles du développement, atteintes à la santé physique et mentale. C’est un choix de société qui est en jeu. Sommes nous prêts à accepter que des enfants dorment dehors alors que la République est fondée sur des principes de solidarité et de dignité ? Sommes nous prêts à fermer les yeux sur la détresse de celles et ceux que nous devrions protéger en priorité ? Il est de notre responsabilité collective de refuser cette fatalité et d’agir avec détermination pour que chaque enfant ait un toit et un habitat digne. loi de finances pour 2024, notre collègue Mathilde Ollivier avait défendu, contre l’avis du Gouvernement, un amendement visant à créer 6 000 places supplémentaires d’hébergement d’urgence. Nous l’avions voté. C’était alors un message fort envoyé par le Sénat. Malheureusement, cet amendement avait finalement été supprimé. Mais, disons le clairement, la simple multiplication des places d’urgence ne résoudra pas structurellement la crise du logement. Le Gouvernement, malgré des discours empreints de compassion, a entériné en 2025 un budgétaire qui rend impossible l’objectif « zéro enfant à la rue proclamé dès 2022. Maintenir les 203 000 places d’hébergement existantes en 2024, sans augmentation significative, revient à abandonner des milliers d’enfants à la précarité. le Gouvernement n’est pas le seul responsable. Osons le dire : certaines municipalités, mues par des considérations idéologiques, refusent obstinément de construire les logements sociaux nécessaires. Ces blocages locaux accentuent les inégalités territoriales et aggravent la saturation des dispositifs d’hébergement. Refuser de construire des logements sociaux, c’est condamner des familles entières à l’exclusion. C’est aussi faire peser sur la société et les associations une charge qui devrait incomber aux pouvoirs publics. Ces derniers mois, ce sont des initiatives associatives et citoyennes qui ont pallié les défaillances de l’État,

Ce n’est qu’en offrant une solution pérenne que nous pourrons briser le cycle de l’exclusion. Cela passe par la mise en œuvre effective du plan Logement d’abord 2. Ce plan, s’il était correctement financé et accompagné d’une programmation pluriannuelle ambitieuse, permettrait de garantir un accès durable au logement pour les familles vulnérables. Il est temps d’accélérer la transformation qualitative du parc d’hébergement. Il faut sortir définitivement de la logique des nuitées hôtelières, trop coûteuses et inadaptées aux besoins des familles, et investir dans des solutions d’accueil dignes et durables. Nous devons également renforcer les dispositifs d’accompagnement global afin de garantir une insertion sociale et professionnelle pérenne pour ces familles. Nous ne pouvons plus accepter que des enfants, nos enfants, soient laissés au bord du chemin. Il est temps de transformer les promesses en actes. Il est temps d’affirmer, par des mesures concrètes et des moyens à la hauteur, que la France ne tolérera plus qu’un seul enfant dorme dehors. En 1948, la Déclaration universelle des droits de l’homme proclamait que « toute personne a droit à un niveau de vie suffisant

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous sommes réunis dans cet hémicycle pour examiner une proposition de résolution visant à mettre fin au sans abrisme des enfants. Nous sommes en 2025, et c’est la honte.

Je souhaite rendre hommage à l’ensemble des acteurs associatifs, aux maires et aux élus locaux qui se démènent au quotidien pour essayer de trouver des solutions. Selon ce baromètre, à la à la veille de la rentrée scolaire 2024, 2 043 enfants se trouvaient sans solution d’hébergement, soit une hausse de 120 % par rapport à 2020. Sur ces plus de 2 000 enfants à la rue, 467 ont moins de 3 ans ! Ces chiffres ne sont pas exhaustifs puisque les personnes sans abri ne font pas forcément appel au 115 ou, pire, n’arrivent pas à joindre ce numéro d’urgence.

« apporter un toit à toutes celles et à tous ceux qui sont aujourd’hui sans abri ». Nous ne pouvons que constater l’échec de cet engagement. De multiples facteurs, au delà de l’inefficacité de l’action politique des gouvernements depuis 2017 – j’y reviendrai –, expliquent

même temps, les loyers du parc privé ont augmenté de 56 % en vingt ans et sont devenus inaccessibles pour de nombreux foyers. La crise de la construction entraîne

J’en viens maintenant à l’action des différents gouvernements depuis 2017 contre le sans abrisme. Le bilan relatif à la lutte contre le mal logement et la perte de logement n’est pas bon. À l’occasion de l’élection présidentielle de 2022, la Fondation pour le logement des défavorisés soulignait que le logement n’avait jamais été une priorité depuis 2017.

à la solidarité et au renouvellement urbains). Le fond de l’air est mauvais et, sous la pression de l’extrême droite, je crains un abandon des principes fondamentaux et juridiques de l’accueil qui ne permettent même plus de protéger des femmes enceintes et des enfants de moins de 3 ans. Notre groupe est mobilisé depuis de nombreuses années pour tenter de faire reculer le sans abrisme. Un travail de fond s’est ainsi engagé avec l’adoption le 24 janvier 2024 de la proposition de loi de notre collègue Rémi Féraud et du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain visant à mettre en place un décompte annuel des personnes sans abri dans chaque commune. La première étape nécessaire à l’élaboration d’une réelle politique de mise à l’abri des personnes à la rue, à la prévention des situations de grande exclusion et à l’insertion durable des publics concernés consiste en effet à recenser précisément les besoins dans toutes nos communes, en particulier dans le milieu rural, où des enfants sont aussi sans toit et sans visibilité.

Ce rapport constate le doublement des personnes sans abri en France, en dix ans : 330 000 en 2024, dont près de 120 000 femmes. Parmi elles, chaque soir, 3 000 femmes et autant d’enfants passent la nuit dehors. Ce rapport émet 22 recommandations importantes que le Gouvernement doit maintenant faire siennes. Je retiens, entre autres, la recommandation n° 2, qui tend à attribuer à l’État la responsabilité de l’hébergement des femmes enceintes et des mères isolées avec un enfant de moins de 3 ans.

pour tous les enfants sans domicile, afin de garantir notamment leur inscription scolaire sans exigence d’un justificatif de domicile. Je veux ici rendre hommage aux personnels de l’éducation nationale qui veillent à accueillir inconditionnellement tous les enfants, en particulier ceux qui sont confrontés à des conditions d’existence très difficiles. En raison de l’urgence de la situation, les sénateurs socialistes voteront avec conviction la proposition de résolution que nous examinons aujourd’hui. Nous souscrivons aux mesures proposées, dont le principe du logement d’abord, en garantissant un hébergement inconditionnel inconditionnel aux personnes en situation de détresse, et l’adoption d’une loi de programmation pour l’hébergement et le logement, en portant une attention particulière aux enfants et aux familles.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je remercie tout d’abord mes collègues qui ont tenu à mettre en lumière ce sujet si grave. Dans le Maine et Loire, le nombre d’enfants à la rue a diminué de 50 % entre 2023 et 2024. C’est encourageant, mais c’est encore À l’échelle nationale, en revanche, leur nombre a augmenté de 120 % depuis 2020. Nous sommes malheureusement encore loin de l’objectif promis de « zéro enfant à la rue

ils ne prennent en considération que les appels au 115. Ils ne tiennent pas non plus compte de tous ceux qui vivent dans des abris tels que des squats ou des logements insalubres ou surpeuplés. Les conséquences du sans abrisme sont terribles, pour tous, adultes comme enfants. Mais, pour ces derniers, il revêt un caractère particulièrement injuste et révoltant, car il les prive d’un environnement sûr et stable, pilier indispensable à leur équilibre. Un enfant sans abri, ce n’est pas qu’un problème de logement. Le sans abrisme des enfants a des répercussions sur leur présent et sur leur avenir. Il met en danger leur santé physique autant que mentale, ainsi que leurs capacités d’apprentissage, et compromet sérieusement leurs chances de réussite scolaire. L’absence de domiciliation peut rendre plus difficile l’inscription même à l’école. Un enfant devrait vivre le présent avec insouciance et rêver de son avenir, et non lutter chaque jour pour le lendemain. Un enfant qui vit dans la rue, c’est l’échec d’une responsabilité collective : celle de l’État, celle des départements et celle des parents. N’ayons pas peur des mots : faire vivre son enfant dans la rue, c’est de la maltraitance, même involontaire. Pourtant, le nombre d’hébergements d’urgence n’a jamais été aussi élevé. Mais ces solutions seront toujours insuffisantes, car le nombre de personnes sans abri augmente lui aussi. Et elles ne sont, par définition, que temporaires. Malgré tout, à titre personnel, je pense qu’il faut continuer de proposer davantage de places d’hébergement d’urgence,

Une fois que l’on a dit cela se pose la question des financements. Certains départements sont déjà à bout de souffle : ils ne peuvent pas faire davantage, alors qu’ils doivent déjà opérer des choix difficiles pour l’accomplissement de l’intégralité de leurs missions. Sur ce sujet comme sur beaucoup d’autres, le Gouvernement doit donc agir en concertation avec eux. Il faut des logements pérennes. Les enfants et leurs familles doivent avoir un toit, une vie normale.

Pour ce qui est du logement social, comment ne pas être tenté de prendre le problème dans l’autre sens, quand on sait que 70 % des ménages français y seraient éligibles ?

On constate que la socialisation accrue du parc immobilier est peut être l’une des causes du problème, puisqu’elle conduit à une pénurie de logements pour celles et ceux qui en ont réellement besoin.

Parce que le moindre enfant qui grandit dans la rue représente à lui seul une situation inacceptable, le groupe Les Indépendants soutiendra cette proposition de résolution.

Car, s’il est une évidence, c’est bien celle que nous ne pouvons pas laisser se développer la misère que l’on observe encore bien trop souvent dans notre pays, quand elle frappe les enfants.

Face à des besoins croissants en matière d’hébergement, je reste convaincue que seule une coopération renforcée entre associations, collectivités territoriales et État permettra d’apporter des réponses concrètes et durables. Je le dis, non pas pour me défausser, mais parce que, dans une période

grâce à l’essor des attributions de logements sociaux, à la création de places en intermédiation locative et au renforcement de l’accompagnement social. Si l’objectif premier est d’accélérer les sorties vers le logement pérenne, il est aussi indispensable de développer des solutions d’hébergement pour ne laisser aucun enfant grandir à la rue ou dans un état de précarité préjudiciable à sa santé, à son éducation et, plus globalement, à son développement. Aussi, le deuxième axe de l’action du Gouvernement consiste à garantir la mise à l’abri inconditionnelle des personnes grâce à un parc d’hébergement suffisamment étendu

L’objectif du deuxième plan Logement d’abord est de consolider encore davantage leur place dans l’accompagnement des personnes à la rue et, notamment, des familles. La dernière période hivernale a fait l’objet d’une attention toute particulière. L’instruction ministérielle du 5 novembre 2024, que j’ai signée, a renforcé l’action des services de l’État en période de grand froid, en prévoyant l’élargissement des horaires des accueils de jour, l’ouverture de centres d’accueil nocturnes exceptionnels et l’intensification des maraudes pour offrir boissons chaudes, couvertures et solutions d’hébergement. À partir du 1 novembre, cette mobilisation exceptionnelle a permis aux préfets d’activer vingt huit plans Grand froid, de renforcer les dispositifs dans cinquante six départements et d’ouvrir près de 2 000 places supplémentaires.

de créer dans les prochains mois 2 000 places d’hébergement spécialisé pour les femmes victimes de violences ou à la rue avec leurs enfants, qui viendront ainsi compléter les 11 000 places existantes, ainsi que les 2 500 places pour les femmes sortant de maternité avec leurs bébés. Ces places spécialisées ont un coût à la place plus élevé que les autres, car elles impliquent un accompagnement social plus qualitatif, notamment des enfants.

doté de 10,3 millions d’euros en 2025, a été mis en place pour réaliser des travaux d’amélioration du bâti et adapter les logements aux besoins des enfants et des familles, notamment par la création d’espaces partagés, de cuisines, ou encore d’espaces de jeu. En outre, je tiens à insister sur le fait que l’accès à l’alimentation est un enjeu primordial pour améliorer les conditions de vie, notamment des ménages hébergés à l’hôtel.

à une alimentation saine et variée. Les mesures déjà mises en œuvre et celles qui sont à venir visent à prévenir l’exposition des enfants aux situations de précarité,

dans les familles avec enfants, est au cœur du dispositif « Un chez soi d’abord », qui, expérimenté depuis 2011, a prouvé toute son efficacité pour répondre concrètement à ces besoins spécifiques de prise en charge. Je travaille en lien étroit

Ses conclusions conduiront à la consolidation des axes de la politique structurelle que j’entends mener pour lutter contre le sans abrisme. Mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement poursuit son action